je vous remercie

que ce projet de loi prévoit, sans étude d'impact, sans concertation avec les parties prenantes et sans véritable évaluation, de modifier la qualité des rapports locatifs telle qu'elle est définie par la loi de 1989. Cet article propose de modifier les règles relatives à la révision des loyers en zone tendue et la contribution du locataire à la suite de la réalisation de travaux, tout cela dans un temps d'examen parlementaire extrêmement contraint.

puisse avoir lieu avant que le Parlement, qui bien évidemment doit garder son pouvoir d'appréciation, soit saisi des modifications proposées ». Si l'objectif du conditionnement de l'augmentation des loyers à la réalisation des travaux

connaissons toujours un mouvement global de hausse des loyers, due à une spéculation foncière et immobilière dont nous ne sommes pas près de sortir. En outre, encore une fois, nous ne disposons d'aucun élément relatif aux moyens financiers que le Gouvernement compte déployer pour accompagner cette réforme. Or il faudrait mobiliser des ressources financières abondantes, d'accès facilité pour le plus grand nombre, au coût par conséquent le plus réduit possible ; cela ne semble pas à l'ordre du jour ... La parole

Il ne me semble pas opportun d'introduire ces dérogations, qui ne sont pas justifiées pour ce dispositif- lequel ne concerne que les évolutions de loyer et le partage des économies de charges -, ni de retarder l'entrée en vigueur de ces dispositions. Tel est le sens de cet amendement. L'amendement

La commission a en outre estimé qu'il est légitime d'exercer une pression particulière sur les bailleurs dont les loyers peuvent continuer de progresser par indexation mais selon un calendrier cohérent avec l'article 3 , ce qui ne permet pas de retenir la date de 2021 et qui explique le choix de 2024 pour appliquer le conditionnement des hausses de loyer

qu'un propriétaire occupant. Elle a donc appliqué, par souci de cohérence, le dispositif proposé par le Gouvernement à l'article 3 du projet de loi. Par ailleurs, la date de 2033 s'applique aux copropriétés connaissant de graves défaillances

Le Haut Conseil pour le climat a ainsi dénoncé, dans son rapport remis au Premier ministre, la faiblesse des mesures proposées par le Gouvernement pour se conformer à la transition énergétique. De même, le dernier rapport du GIEC a enjoint aux États d'inverser la tendance d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, sous peine d'assister aux effets irréversibles de cette pollution, sur notre planète et pour l'humanité. Face à ces nombreux constats, il est urgent de faire évoluer les mentalités et la manière de consommer. Des écogestes simples et quotidiens permettraient de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons repenser nos pratiques énergétiques et faire preuve de frugalité en la matière. Ainsi, c'est un non-sens économique, écologique et énergétique que de continuer à chauffer des locaux lorsque ceux-ci ne sont pas occupés. Tel est donc le sens de cet amendement qui vient instaurer une sobriété énergétique en dehors des heures d'activité au sein des bâtiments non résidentiels. Une bonne isolation évite en effet le refroidissement des murs et diminue donc la condensation intérieure. Les locaux bien isolés concentrent suffisamment de chaleur pour que les coupures de chauffage puissent être effectuées lorsque les pièces à vivre ne sont pas occupées. Ce geste permettrait une économie évaluée entre 22 % et 26 % par rapport à un fonctionnement constant du système de chauffage. Enfin, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, régler la température à 19 degrés dans les pièces à vivre serait bénéfique pour la santé des travailleurs et permettrait la diminution de la consommation énergétique de 7 %.

Un bâtiment bien isolé et chauffé en période d'activité retient suffisamment de chaleur pour que des économies d'énergie puissent être faites lorsque les locaux ne sont pas occupés. La mesure proposée permettrait également de réaliser des économies financières, du fait d'une moindre consommation énergétique.

les périodes d'inoccupation des locaux d'une durée égale ou supérieure à 24 heures consécutives, la température moyenne du chauffage est limitée à 16 degrés et à 8 degrés au-delà de 48 heures.

Outre la remise à plat de ces aides, annoncée par le Gouvernement, il demeure indispensable d'accompagner les ménages, afin de les inciter à engager rapidement des travaux qui leur bénéficieront directement, soit sur leur facture énergétique, pour les occupants, soit sur la valeur de leur bien, pour les propriétaires bailleurs. Le présent amendement vise à instaurer un référent chargé de les accompagner. Désigné au sein des EPCI compétents en matière d'habitat, ou à défaut dans les communes, il les informera des travaux possibles, ainsi que des aides publiques mobilisables. Quel est l'avis de la commission ?

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale s'engagent avec plus de force dans la lutte contre l'habitat indigne, et certaines d'entre elles se sont saisies de la possibilité offerte par la loi ALUR d'instaurer un permis de louer dans certains secteurs géographiques. Or, dans l'habitat dégradé, nous rencontrons souvent des logements excessivement énergivores. Le permis de louer pourrait dès lors trouver toute son utilité pour accélérer la rénovation énergétique des logements classés F et G. Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités locales ayant institué ce dispositif de refuser l'autorisation lorsque le logement constitue une passoire énergétique.

la performance énergétique des logements est d'ores et déjà incluse dans les critères d'attribution d'un permis de louer, car non seulement le bailleur doit préciser dans le formulaire de demande la consistance du logement, conformément au décret « décence », mais aussi, pour obtenir le permis, il doit transmettre

Sans modifier les critères de décence, nous considérons que le bailleur mettant en location un bien immobilier classé F ou G au regard du diagnostic de performance énergétique doit être incité à le rénover. rénover. Par cet amendement, il s'agit d'accélérer la rénovation des logements du parc locatif privé, en supprimant le bénéfice du tiers payant des APL pour les propriétaires qui proposent à la location des passoires énergétiques. Je tiens à le préciser, il ne s'agit pas de la suppression du bénéfice de l'APL pour le locataire. Afin de mettre en oeuvre cette mesure, il est également proposé que le bailleur transmette aux CAF le contrat de location, assorti du diagnostic de performance énergétique. C'est à cette condition qu'il pourra bénéficier du tiers payant. La parole est à Mme Angèle Préville,

des travaux de rénovation thermique des logements en vue d'améliorer le confort thermique des locataires. On le sait, les propriétaires bailleurs sont aujourd'hui

est à Mme la ministre. Comme vous le rappelez, l'article 140 de la loi ÉLAN permet aux collectivités volontaires d'engager une nouvelle mesure d'encadrement des loyers dans le cadre d'une expérimentation. Celle-ci a été ouverte pour une durée de cinq ans. Comme vous le savez, elle est mise en oeuvre depuis le 1 juillet

est à Mme la ministre. L'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit déjà qu'une contribution pour le partage des économies de charges ne peut être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. Le seuil de performance énergétique défini par l'arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social est déjà plus ambitieux que le seuil de 331 kilowattheures par mètre carré et par an défini à l'article 3 .

la commission ? L'argumentation du Gouvernement est surprenante, car elle devrait s'appliquer de la même manière à la contribution des locataires à la suite de travaux d'économie d'énergie dans le parc privé, visée à l'article 3 , et que le Gouvernement a approuvé à l'Assemblée nationale et, à l'instant même, devant notre assemblée. La commission a ajouté cet article 3 pour maintenir le parallélisme des deux dispositifs, dans le parc privé et dans le parc social,

qui figure déjà dans les DPE délivrés au vu de la réglementation en vigueur, et de supprimer la double étiquette en énergie primaire et finale pour la classification du bâtiment en fonction des valeurs de référence, donc les étiquettes A à G, ainsi que la mention des dépenses d'énergie réelles du dernier occupant. Une double étiquette sur la consommation en énergie du bien en énergie primaire et en énergie finale risquerait en effet de créer beaucoup de confusion chez les particuliers. Pour un DPE d'un logement chauffé au gaz, les deux étiquettes seraient identiques, contrairement à l'électricité où elles seraient très différentes, sans que l'explication de cet écart soit directement compréhensible pour le ménage. Pour les dépenses réelles d'énergie, il sera souvent très difficile, pour le bailleur, d'obtenir des informations de la part du locataire, ce qui rendrait l'obligation impossible à respecter.

le DPE. Il est vrai que l'affichage des dépenses réelles pose des difficultés d'application pratiques et dépend des habitudes de consommation ou de la composition du foyer.

Pour prévoir ces épisodes amenés à durer, le bâti devra lui aussi faire preuve d'adaptation et de résilience. C'est ce que nous proposons au travers de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ?

du 1 janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives

pour présenter l'amendement n° 31 rectifié. Le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation d'énergie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec 7,4 millions de passoires énergétiques dans notre pays, il est évident que la rénovation énergétique constitue la condition pour atteindre nos objectifs en la matière, ainsi que l'espoir d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Or le projet de loi se contente de consacrer l'obligation pour les bâtiments à usage d'habitation de ne pas excéder le seuil de 330 par mètre carré et par an de consommation d'énergie primaire, soit les classes F et G, en 2028. Il ne prévoit aucune sanction. Qu'il faille inciter les propriétaires plutôt que les contraindre, nous le concevons. Ce sera le cas, d'après le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances. Nous proposons d'ailleurs d'avancer l'entrée en vigueur des mesures mesures incitatives : mention de l'obligation de performance énergétique dans les annonces immobilières, les actes de vente et les baux. En effet, il convient d'informer nos concitoyens dans les meilleurs délais. Mais l'incitation ne sera pas suffisante, notamment lorsque le propriétaire n'est pas l'occupant, puisqu'il ne règle pas la facture d'énergie pour son bien énergivore à la fin du mois. Ce sont donc les locataires qui sont financièrement pénalisés et qui continuent d'avoir froid l'hiver et chaud l'été. Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques dans le marché locatif, de manière progressive et raisonnable. En 2022 : fin de la location des biens immobiliers classés G ; nous aurons au moins un objectif atteint à la fin du quinquennat, car il est bien trop facile de fixer des objectifs pour le prochain, de même qu'il est bien trop facile de laisser les générations futures régler l'urgence climatique.

aux défis du dérèglement climatique. Mes chers collègues, le dispositif proposé n'inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant ni les biens vendus. Il fixe ainsi un calendrier réaliste, certes moins ambitieux que le programme du Président de la République alors candidat rénovation de la moitié des logements-passoires dès 2022 et interdiction de la location des passoires énergétiques à compter de 2025. Un fonds public était prévu pour prendre intégralement en charge les travaux des propriétaires les plus précaires.

l'amendement n° 301 rectifié. Dans notre pays, on compte encore 7,4 millions de passoires énergétiques, c'est-à-dire des logements classés F et G, alors que le secteur du bâtiment représente 45 % de la consommation de l'énergie et 20 % des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique constitue donc l'un des principaux leviers de la transition écologique et de l'atteinte des objectifs ambitieux que le projet de loi entend fixer.

permettant d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. Le présent amendement vise à accélérer le rythme de réhabilitation des passoires énergétiques ; n'oublions pas que c'est une nécessité pour nos concitoyens aux revenus modestes qui sont locataires dans des passoires énergétiques. Il tend à instaurer un objectif intermédiaire la fin de la location des biens immobiliers classés G en 2022. Nous affirmons clairement l'interdiction de la location de l'ensemble des passoires énergétiques en 2028. Cela ne signifie pas la fin de ces dernières, puisque le dispositif n'inclut ni les biens pour lesquels le propriétaire est occupant ni les biens vendus. La parole

de limiter le dispositif aux zones tendues dans lesquelles les propriétaires perçoivent des loyers suffisamment élevés pour faire face aux travaux de rénovation.

Par ailleurs, avancer d'une année l'obligation d'affichage de la non-conformité future des passoires énergétiques sera un signal permettant aux propriétaires d'anticiper bien avant 2028 les travaux à réaliser. Quel

soutenons donc le principe d'une forme d'interdiction pour les logements les plus énergivores au sein de la classe G à travers des critères de décence. Pour le reste des logements classés F et G, il semble préférable de travailler à la mise en place de dispositifs opérationnels contribuant ou incitant à la rénovation des passoires énergétiques plutôt que d'inscrire une date butoir dans la loi.

est à Mme la ministre. Le présent amendement cible le champ d'application des dispositions sur l'affichage des charges dues à la consommation énergétique sur les biens immobiliers résidentiels.

supprimer la mention des dépenses réelles du dernier occupant et à instaurer une sanction administrative pour les manquements à l'obligation de mentionner le classement du bien. Quel est l'avis de la commission ? classement du bien. Quel est l'avis de la commission ? Par cet amendement, le Gouvernement corrige la rédaction qu'il avait proposée à l'Assemblée nationale en plusieurs points. Il précise le contenu de l'audit énergétique en retenant non plus un haut niveau de performance énergétique, mais le fait d'atteindre l'étiquette E, en prévoyant la présentation de travaux avec un coût chiffré en supprimant l'obligation de simulation qui figurera dans l'arrêté. Il supprime en outre la mention des dépenses énergétiques réelles. Enfin, il crée une sanction administrative. La commission a approuvé l'ensemble de ces évolutions. L'avis est donc favorable.

Il crée une norme maximale de consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation applicable à partir du 1 janvier 2028, des mesures coercitives être pouvant être prise en 2023 lors de l'examen de la loi quinquennale prévue à l'article 1 A. Toutefois, alors que le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et 25 % des émissions de gaz à effet de serre, j'ai tendance à considérer une obligation de rénovation des passoires thermiques dépourvue de sanction comme un voeu pieux n'en garantissant aucunement une réelle application. C'est

Le secteur du bâtiment, qui pèse 10 % de notre produit intérieur brut et représente plus d'un million d'emplois, doit impérativement s'inscrire dans une dynamique de développement durable, y compris sur le plan économique. Réglementer et transformer les pratiques locatives, c'est envoyer un signal fort aux 390 000 entreprises françaises du bâtiment, afin d'encourager l'innovation en faveur de matériaux et de solutions constructives. C'est aussi redynamiser la filière pour rénover mieux. Sur le plan social, c'est sortir 5,1 millions de ménages du froid et de charges locatives insoutenables. Sur le plan environnemental, c'est acter l'urgence climatique en s'attaquant aux secteurs des plus énergivores. Certes, chacun ici rappelle qu'il faut instaurer une obligation de rénovation des passoires thermiques, celles-ci constituant une aberration, et brandit son triptyque : incitation, obligation, contrainte. Mais dès qu'il s'agit de l'appliquer effectivement, il n'y a plus de véritable solution. La définition d'une sanction est reportée à 2028. Cela rend douteuse la perspective que ces rénovations puissent effectivement voir le jour. Pour notre part, nous souhaitons réaffirmer l'urgence à laquelle nous sommes confrontés et les risques de non-aboutissement qu'induit le report à une prochaine mandature. Par cet amendement, nous entendons donc sécuriser le principe de sanctions, en veillant à ce que leur définition ait lieu durant ce quinquennat. La

Le scrutin est ouvert.

Le Sénat n'a pas adopté. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription de la suite du projet de loi relatif à l'énergie et au climat à l'ordre du jour du vendredi 19 juillet, le matin et l'après-midi.

est ainsi libellé : La parole est à M. Éric Gold. La réalisation d'un audit énergétique obligatoire pour les passoires énergétiques peut constituer un outil incitatif intéressant, à condition de s'en emparer pour informer au mieux nos concitoyens des avantages à rénover le bâti. Le présent amendement vise à mentionner à titre indicatif l'impact des travaux proposés par l'audit sur la facture énergétique. Si l'investissement initial peut sembler prohibitif et rédhibitoire, il convient de démontrer qu'il sera rentabilisé par les économies d'énergie. Quel est l'avis de la commission ?

De surcroît, outre les aides nationales, nombreuses sont les collectivités qui proposent des aides locales et leurs conditions d'attribution varient d'un territoire à l'autre. Dès lors, il est intéressant de personnaliser davantage l'audit énergétique en mentionnant les conditions d'attribution des aides destinées aux travaux de rénovation énergétique. Quel est l'avis de la commission

en vue d'inciter les propriétaires à rénover leurs biens immobiliers classés F ou G en améliorant la connaissance de ces derniers : obligation de réaliser un audit énergétique pour ces logements ; mention du classement du bien et du montant des dépenses énumérées dans le diagnostic de performance énergétique dans les annonces de vente et de location, ainsi que dans les contrats de location. Ces mesures ne sont pas contraignantes et il est peu compréhensible de reporter leur application au 1 janvier 2022 au regard de l'urgence climatique. Mes chers collègues, nous pouvons mettre en oeuvre ces mesures sans tarder pour espérer qu'une dynamique s'engage rapidement dans la rénovation du bâti. Autrement, je le répète, les objectifs de la politique énergétique ne seront pas respectés. Par cet amendement, nous vous proposons d'avancer l'entrée en vigueur de ces mesures à un an après la publication de la loi.

De même, il faudra définir ce qu'on attend de l'audit énergétique et les conditions dans lesquelles les informations seront fournies. Il faut laisser le temps que tout cela se fasse et soit intégré par les professionnels. Avis défavorable.

énergétiques donnent lieu à des travaux et à des documents approfondis qui ne peuvent être aisément résumés. Cela représenterait donc une masse très importante de documents qui ne seraient pas exploitables. Il ne semble pas envisageable d'exiger une synthèse numérique aisément exploitable de manière informatisée et statistique, sauf à renchérir de manière substantielle le coût des audits, ce qui serait contradictoire avec la volonté d'accroître le recours à cet outil, en particulier pour les passoires énergétiques. Il est donc proposé de supprimer la transmission pour les seuls audits énergétiques,

L'élaboration de ces parcours permet la personnalisation des travaux proposés et une planification de ces derniers par étapes en vue d'aboutir à une rénovation complète, et donc plus efficace des logements. La priorité doit être d'accompagner les ménages en situation de précarité énergétique durant toute la durée de la rénovation de leur logement. Le présent amendement vise donc à préciser dans les missions de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, que la lutte contre la précarité énergétique doit être réalisée dans le cadre d'un tel parcours.

à adopter le parcours énergétique de manière systématique. Il convient plutôt, selon moi, de laisser l'agence adapter ses modes d'action aux publics et aux objectifs recherchés. Avis défavorable.

indigents du fait de leur consommation énergétique, ou encore les révisions de loyer. Les informations listées ne font actuellement pas l'objet d'un suivi quantitatif. Il ne semble pas envisageable de le permettre en prévoyant des obligations déclaratives pour les ménages et les entreprises, cela ferait peser une charge administrative démesurée sur des millions de nos concitoyens. Un observatoire est en cours de mise en place et il s'attachera à examiner les moyens permettant de disposer des meilleures informations possible. En l'état, il me semble prématuré de s'engager sur une liste aussi précise d'informations chiffrées.

le CGEDD, dans leur rapport d'avril 2017, de pallier cette lacune en créant un observatoire pour disposer enfin des éléments nécessaires au pilotage de la politique de rénovation énergétique. Ne pouvant créer un observatoire par voie d'amendement, la commission avait donc

qui ne devraient pas poser de problème ! La transition écologique ne se fera pas avec partiellement. Ouvrir la voie vers un modèle de société viable appelle à créer un système cohérent qui englobe l'ensemble de nos activités économiques. Les investissements financiers en font pleinement partie ils constituent un levier décisif qu'il convient de contrôler afin d'acter la réorientation de notre économie vers un fonctionnement durable. À cet égard, certaines expertises tentent d'ouvrir la voie aux démarches nécessaires à cet objectif. Dans ses recommandations sur les projets de plans nationaux énergie-climat des États membres, la Commission européenne énonce clairement que la France doit faire preuve de transparence sur ses subventions aux énergies fossiles tout en prenant des mesures pour y mettre fin.

Une telle situation est inacceptable, surtout après le vote intervenu hier soir. Nous ne pouvons pas réguler à domicile s'il s'agit de cautionner des projets écocides à l'étranger, en l'occurrence avec de l'argent public. En 2015, ce paradoxe gênant était déjà mis sur la table. L'État s'engageait à mettre fin aux garanties à l'export s'agissant des centrales à charbon. Aujourd'hui, alors que limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici à la fin du siècle nous appelle à laisser dans le sol plus de 80 % des réserves de charbon, un tiers des réserves de pétrole et la moitié de nos réserves de gaz, nous souhaitons que la France se conforme à ses engagements internationaux et qu'il soit mis fin à ces subventions en faveur des énergies fossiles

Le Gouvernement a déjà annoncé son intention de mettre fin aux garanties à l'export en soutien de la production de charbon dans la prochaine loi de finances. L'amendement n° 279 sera donc satisfait sur ce point. Pour le reste, je ne vois pas ce que nous aurions à gagner à avoir le bilan complet des garanties déjà octroyées. Quant aux pistes d'action pour mettre fin aux garanties à une échelle plus grande que la France, elles passent bien davantage par des négociations dans un cadre européen ou multilatéral que par la production d'un rapport. Enfin, s'agissant de l'interdiction de toutes les garanties à l'export, n'oublions jamais que si elle était appliquée unilatéralement, elle aurait pour effet d'évincer les entreprises françaises des marchés internationaux. C'est pourquoi la commission est défavorable à ces deux amendements.

et de mesurer l'impact d'une éventuelle réduction de ce soutien sur chaque type d'énergie. Un rapport est prévu à l'article 3 . Par ailleurs, comme l'a souligné M. le rapporteur,

qu'il fallait mobiliser l'État, les collectivités, les entreprises privées et le système bancaire. Très bien,

2019 s'élève à 11 milliards d'euros. Ces sommes freinent l'essor de la transition écologique en avantageant les secteurs polluants et sont perdues pour le budget de l'État, alors entre autres, des projets de transition écologique et à accompagner les ménages et certains secteurs d'activité. À ces exonérations et taux réduits, il faut ajouter les subventions en faveur des énergies fossiles sous forme de garanties à l'export, délivrées par Bpifrance pour le compte de l'État. Or, pour accélérer la transition écologique et être cohérent avec l'accord de Paris, il est temps d'envoyer un message fort : les énergies fossiles polluent et doivent rester dans le sol. C'est un non-sens de continuer à subventionner leur utilisation. La France, pays hôte du G7 en 2019, s'est engagée à supprimer les subventions aux énergies fossiles d'ici à 2025. Elle s'est dotée d'un objectif de réduction de la consommation de 30 en 2030 dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et propose dans ce projet de loi de le renforcer, en Il faut maintenant que cet engagement soit suivi d'actions dans notre pays pour éviter que ces objectifs ne restent des voeux pieux. Ces informations devront notamment figurer dans l'annexe au projet de loi de finances. Il s'agit également de trouver des solutions avec les secteurs concernés pour permettre une suppression progressive des subventions, afin de maîtriser les effets sur l'emploi et la compétitivité des entreprises.

Je rappelle aussi que, s'agissant du territoire national, la loi Hydrocarbures a déjà prévu l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures en 2040. Enfin, ne jouons pas aux pompiers pyromanes : le rapport demande la fin des subventions mais, dans le même temps, s'inquiète des conséquences sociales.

vise à remettre au Parlement un rapport relatif aux incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique. J'ai eu l'occasion de l'indiquer, une mission de l'Inspection générale des finances et du

Ces bilans me semblent importants pour permettre aux acteurs concernés d'identifier les leviers de réduction de leurs émissions et pour informer le public. Cet amendement vise donc à réintroduire les dispositions supprimées, en y apportant quelques ajustements allant dans le sens d'une simplification. Il tend d'abord à préciser le contenu du plan de transition prévu, avec la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs concernés et une rédaction simplifiée. Il prévoit ensuite une augmentation limitée du montant maximal de la sanction, qui reste cependant suffisant pour assurer son caractère incitatif. Il comporte un ajout pour dispenser les entreprises soumises au reporting extrafinancier de l'élaboration du plan de transition prévu et des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, un dernier ajout vise à permettre aux collectivités d'être exonérées de la réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre

des modalités simplifiées de mesure des émissions. À ma connaissance, cet alinéa est resté pour l'instant lettre morte, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous sommes en tout cas bien d'accord, sans la mobilisation des territoires, nous ne tiendrons pas nos objectifs.

Au total, je constate que la principale raison ayant motivé la suppression du dispositif en commission n'a pas disparu. En effet, par rapport au droit existant, l'amende serait multipliée par plus de dix dans le premier cas, et plus de trente dans le second. Or ce montant n'est cohérent ni avec le montant des contraventions applicables en droit pénal ni avec le coût de production du bilan. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la lecture du rapport remis au Président de la République en 2015 sur l'ordonnance ayant créé cette sanction : « Il est

s'agit, là aussi, de rétablir une avancée : l'Assemblée nationale avait introduit une obligation de reporting des acteurs financiers sur les risques de l'investissement en matière de durabilité.

sur le type d'informations que les institutions financières auront à fournir dans le cadre de leur reporting sur la prise en compte des risques de leurs investissements en matière de lutte contre le changement climatique. Ces risques sont d'une double nature : il y a ceux liés à l'investissement lui-même,

l'importance de cet acteur. M. Fink disait dans, lundi dernier : « Notre responsabilité est de guider nos clients en leur expliquant pourquoi il est pertinent d'investir dans les entreprises qui se préparent au mieux à la prise en compte des enjeux environnementaux, qui se concentrent le mieux sur le développement durable.

la transition énergétique pour la croissance verte, qui a obligé les investisseurs institutionnels à publier un rapport annuel et des informations sur les modalités de prise en compte, dans leur politique d'investissement, des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux,

Il a été constaté, par exemple, que le programme de politique monétaire mis en oeuvre par l'Eurosystème et la Banque centrale européenne, la BCE, ont conduit à la création d'un très important portefeuille d'investissement dans les entreprises européennes : plus de 77 milliards d'euros d'encours, dont 53 milliards pour la Banque de France. Il est donc important que la Banque de France fasse aussi un reporting précis du caractère durable des investissements en vue d'informer l'ensemble de la population. Le sous-amendement n° 459 rectifié vise à faire publier dans la politique des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion une évaluation détaillée et chiffrée des ressources qui sont mises en oeuvre et dédiées aux objectifs de la transition énergétique et écologique. Le sous-amendement n° 460 rectifié prévoit que le rapport annuel et les informations mis à la disposition des souscripteurs par les investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion soient rendus publics, et contiennent des informations détaillées traçables

des risques à long terme par les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, en particulier l'évaluation des risques de transition et des risques physiques associés au réchauffement climatique. Il s'agit de permettre l'évaluation des risques de long terme auxquels ils sont exposés, d'informer sur ces risques afin d'éviter l'apparition de risques systémiques que l'on a déjà connus, tels que la dépréciation massive d'actifs carbone, et qui pourraient être engendrés par des mesures réglementaires de lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, il convient que la prise en compte

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à rétablir, avec quelques précisions, un article introduit à l'Assemblée nationale qui permet de mettre les entreprises françaises à la pointe du reporting environnemental.

similaire. Les amendements n 112 rectifié et 329 visent à rétablir l'article 3, dans une rédaction légèrement différente. Or cet article a été supprimé par la commission pour plusieurs raisons tout à fait justifiées.

Dès lors, les modifications proposées reviendraient à appliquer de manière anticipée le règlement. Or il n'y a pas d'urgence à modifier notre droit, d'autant que les dispositions existantes ont été adoptées voilà peu de temps, à l'occasion de la loi de 2015 relative à la transition énergétique. En second lieu, une partie du dispositif est de nature réglementaire : c'est le cas de la définition des risques physiques et de transition ainsi que de la description de la méthodologie d'analyse, qui figurent actuellement dans la partie réglementaire du code monétaire et financier. Enfin, dans sa rédaction issue de l'amendement n° 112 rectifié, le dispositif fait référence aux risques liés à la biodiversité. Il n'est pas exclu que le Conseil constitutionnel considère que de tels risques ne présentent pas de lien avec le projet de loi en cours d'examen. Pour ce qui concerne les sous-amendements, leur contenu est également problématique. Ils auraient en effet pour conséquence d'apporter davantage de rigidité au dispositif, en étendant son champ d'application, notamment à la Banque de France et aux sociétés d'assurance, et en imposant des obligations nouvelles en termes de méthodologie et d'information. Ces évolutions sont peu utiles au regard du droit existant, puisque les sociétés d'assurances sont déjà incluses dans le périmètre du dispositif et que les obligations de méthodologie et d'information sont détaillées dans la partie réglementaire du code précité. L'avis est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements et sous-amendements.

pourrions aussi évoquer le Fonds de réserve pour les retraites, qui détient des millions d'euros d'obligations dans les entreprises exploitant des mines de charbon en Allemagne et en Afrique du Sud.

de vote. Je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Mme la présidente de la commission des affaires économiques. Il ne s'agit pas de charges supplémentaires et nouvelles pour les entreprises ! Nous parlons ici des investisseurs auxquels les épargnants ou les institutionnels confient leurs fonds.

des grands groupes ... Nous n'avons absolument pas besoin de ce genre de rendez-vous : nous rencontrons toute l'année sur le terrain, avec la délégation aux entreprises, de nombreuses entreprises, généralement d'ailleurs des PME ou des TPE, qui ne cessent de nous dire à quel point le fardeau administratif et normatif

ultérieurement aussi aux autres pays de l'Union. Il est important de donner un signal fort sur le fait que nous souhaitons être en pointe dans ce domaine, et ne pas perdre de temps face à l'urgence.

indiquer la quantité moyenne de CO2 émise par kilomètre et par personne. D'ores et déjà, l'article L. 1431-3 du code des transports oblige toute personne qui ou organise une telle prestation à informer le bénéficiaire de la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Quel est l'avis de la commission ? Les transports concentrant près de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, il est essentiel de mobiliser les professionnels et les consommateurs pour promouvoir la transition énergétique dans ce domaine. Pour autant, le dispositif proposé n'est pas satisfaisant. Tout d'abord, le projet de loi d'orientation des mobilités, en cours d'examen, prévoit en son article 26 AB la nécessité d'assortir les publicités en matière de transport d'un « message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives Par ailleurs, les personnes commercialisant des prestations de transport doivent déjà « fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise », selon l'article L. 1431-1 du code des transports. Ainsi, l'apport du dispositif est limité par rapport au droit en vigueur ou à venir. L'avis est défavorable.

Les propositions qui ont été faites dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités en cours de discussion visent à faire la promotion des mobilités actives : ce n'est pas du tout le même message que celui qui sous-tend évoqué les obligations réglementaires actuelles, monsieur le rapporteur. L'information des donneurs d'ordre en matière de transport ne concerne pas les particuliers.

est à Mme la ministre. Le Gouvernement approuve l'idée d'introduire un critère carbone dans les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, comme le texte en prévoit le principe. Un tel critère est notamment mis en oeuvre dans les appels d'offres pour le solaire photovoltaïque. Toutefois, tous les dispositifs de soutien ne se prêtent pas à l'introduction d'un tel critère. Sa mise en oeuvre peut être excessivement complexe dans certaines situations ou pour certains projets au regard de leur taille. De plus, l'intégration d'un critère carbone peut, dans d'autres situations, ne pas avoir d'impact sur le choix des projets de production lauréats, et donc être inutile en pratique. Le présent amendement vise à répondre à ces deux difficultés en prévoyant de mettre en place des bilans carbone dès lors qu'ils sont techniquement faisables et utiles dans la procédure de sélection. Par ailleurs, les dispositions proposées entreraient en vigueur immédiatement, faisant peser un risque sur l'ensemble des dispositifs de soutien français. Il est prévu de laisser un délai de dix-huit mois permettant de modifier les dispositifs de soutien et de procéder à leur éventuelle validation auprès de la Commission européenne, ce qui nécessite un an. Le sous-amendement

limitations ajoutées. Si le bilan carbone n'est intégré qu'à condition que sa mise en oeuvre soit techniquement possible et qu'elle permette une discrimination effective entre les projets, alors on videra le dispositif d'une partie de sa substance et de son intérêt. Si on ne commence pas par calculer le bilan carbone, on ne parviendra jamais à faire naître des filières plus vertueuses dans notre pays et dans l'Union européenne. Et si aujourd'hui ces filières n'existent pas encore, on constatera que le bilan carbone ne diffère pas selon les projets, mais on en aura au moins connaissance. On nous demande de calculer notre empreinte carbone dans tous les secteurs. Je ne vois pas pourquoi les énergies renouvelables en seraient exonérées, alors que ce sont elles qui doivent être concernées au premier chef. L'avis est favorable, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, qui tend à supprimer les alinéas 1 à 3.

d'une installation de méthanisation. Il est très judicieux d'avoir un bilan carbone pour mettre en place des dispositifs d'aide et de subvention aux projets d'énergie biogaz. Je soutiens donc la rédaction qui a été élaborée par la commission des affaires économiques. Cependant, la rédaction actuelle ne me semble pas suffisamment précise. Il semble utile de nommer, en ce qui concerne la méthanisation, les différents éléments qui concernent non pas l'entretien, l'installation, le transport et le démantèlement de l'unité de production, mais son fonctionnement quotidien, son apport en intrants, la gestion des digestats et sa sécurité, car de nombreux risques pour le bilan carbone y sont associés.

en intrants et de transport des digestats pour leur épandage : il convient de favoriser les projets de méthanisation territorialisés- je l'ai déjà dit -, en cohérence avec les ressources et les possibilités d'épandage du territoire. L'approvisionnement en intrants de proximité, dans des unités de méthanisation avec des tailles cohérentes, paraît donc essentiel. Il faut prendre en compte, ensuite, l'impact des digestats : mal contrôlés, le stockage et l'épandage du digestat peuvent entraîner l'émission de protoxyde d'azote, 300 fois plus impactant sur l'effet de serre que le CO2. Le digestat peut entraîner une perte de carbone organique dans les sols, alors même que ce stockage du carbone organique est envisagé par le Gouvernement

par les fuites des unités de production : à partir de 10 % de fuites, le bilan environnemental serait négatif. Voilà l'explication de cet amendement, qui précise les conditions de la méthanisation.

car c'est un beau sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure, notamment avec la question de la valorisation des boues des stations urbaines et industrielles. Là encore, on va pouvoir trouver de nouvelles valorisations, de nouvelles richesses, à condition que ...

En effet, durant leur stationnement en port, les navires continuent de consommer du carburant polluant et produisent ainsi en continu des particules fines. Diverses études affirment que les émissions de gaz à effet de serre de ces paquebots sont plusieurs milliers de fois plus importantes que celles d'un véhicule terrestre classique. La pollution au fioul lourd tue des milliers de personnes chaque année et les conséquences sur la couche d'ozone sont désastreuses. Les usagers de la route, qui utilisent leur véhicule

économie. Il introduit automatiquement une concurrence entre les ports français et étrangers. En cas d'interdiction générale de tous les navires polluants en France, ces derniers séjourneront tout simplement dans un port voisin, en Italie, en Espagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, et y débarqueront leurs cargaisons qui ensuite circuleront dans le marché intérieur jusqu'aux consommateurs français.

d'une certaine dynamique, et les prix à la consommation, sans pour autant contribuer à diminuer la flotte de navires polluants. Une telle régulation ne peut se faire qu'à l'échelle de l'Union européenne, compte tenu de la proximité géographique entre les ports français et ceux de nos voisins. Imposer unilatéralement une interdiction d'entrée dans nos ports, sans évaluation préalable, sans concertation et sans harmonisation au niveau européen pour un gain environnemental minime, présente bien plus de risques que d'avantages, même si, sur le fond, je partage complètement

à l'environnement et à la santé humaine. Le port de Marseille offre déjà- je sais que vous êtes au courant -des branchements électriques à quai. Il va y investir 20 millions d'euros supplémentaires, d'euros supplémentaires, afin de faire de Marseille le premier port de Méditerranée 100 % électrique d'ici à 2025. Par ailleurs, le schéma national d'orientation pour le déploiement du GNL comme carburant marin prévoit déjà, à l'horizon 2025-2030,